et a ouvert la possibilité aux professionnels de bénéficier d'aide à l'acquisition d'un vélo-cargo. D'autres dispositions ont permis d'amplifier les dispositifs d'accompagnement des ménages dans les ZFE-m.

de leur mobilité. Le montant de l'aide est crucial pour réduire au maximum le reste à charge des ménages, principal frein

comme les transports en commun. Il s'agit donc, vous l'aurez compris, de favoriser les mobilités de substitution, en créant une prime à la mobilité durable dotée de 160 millions d'euros.

qui ne peut être présent ce soir puisqu'il est avec le Président de la République aux États-Unis, véritable événement pour la relation franco-américaine ... Quel veinard ! Le présent amendement prévoit l'affectation d'une partie du fonds vert à la rénovation des sites événementiels afin de les accompagner dans la réalisation des travaux de rénovation thermique et de modernisation de leurs infrastructures. Ces sites participent activement à l'attractivité des territoires. Véritables leviers de dynamisme économique et d'emplois, ils sont également de fabuleuses vitrines à l'international des grands salons et événements qui y sont organisés. Afin d'assurer la modernisation des sites et de leurs structures, un investissement significatif dans la rénovation, notamment thermique, et la gestion énergétique des bâtiments est réclamé et attendu par les professionnels

faire confiance aux territoires : qu'ils déterminent eux-mêmes les meilleurs projets, en cohérence avec leur PCAET

parole est à Mme Martine Filleul. Cet amendement vise à renforcer les crédits prévus pour le financement de l'action dédiée aux voies navigables. Avec 8 500 kilomètres de voies navigables, la France possède le plus long réseau d'Europe, mais elle est aussi l'un de ses plus faibles utilisateurs. En effet, le transport fluvial de marchandises représente moins de 3 % des tonnes-kilomètres transportées. Pourtant, le transport fluvial émet en moyenne cinq fois moins de CO2 à la tonne transportée. est une source d'économie d'énergie extrêmement intéressante, à condition que des investissements soient réalisés sur le réseau. Pour soutenir ce mode de transport, nous proposons de doubler l'enveloppe allouée à Voies navigables de France (VNF) dans le cadre de ce projet de loi de finances, pour atteindre 400 millions d'euros. Cette montée en puissance est indispensable pour moderniser le réseau : rénovation d'ouvrages, restauration de digues ou de berges, automatisation d'écluses, verdissement de la flotte, etc. Elle permettra de

particulièrement enthousiasmante, mais il requiert un investissement au long cours. Cet amendement vise ainsi à lancer un vaste programme d'investissement en la matière permettant, à terme et en partenariat avec VNF, de mobiliser 1 milliard d'euros.

Monsieur le rapporteur

Madame la ministre, lors du débat sur le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, nous étions nombreux sur ces travées à regretter que le développement des réseaux de chaleur n'ait pas été mieux pris en compte dans le texte du Gouvernement. À ce titre, la Cour des comptes a observé que « si la France avait voulu faire de sa politique en faveur des énergies renouvelables (EnR) un levier de lutte contre le réchauffement climatique, elle aurait dû concentrer prioritairement ses efforts sur le secteur des EnR thermiques qui se substituent principalement à des énergies fossiles

la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute de chaleur et de froid ne représentait que 23,4 % en 2020, pour une cible de 34,3 % à 38,9

Depuis 2008, l'État a organisé quatre appels à projets pour contribuer au développement de ces transports en site propre et des pôles multimodaux. Ce dispositif fonctionne et a un levier de levier considérable. : La parole est à M. Hervé Gillé. Nous souhaitons que l'État soutienne les projets de développement et de modernisation des infrastructures et des systèmes de transport urbain. Il a ainsi organisé plusieurs appels à projets pour contribuer au développement des transports en site propre-

Notre amendement vise à instaurer un soutien durable, qui permettra de poursuivre le développement de nouvelles infrastructures de métro, de tramway et de bus à haut niveau de service (BHNS) ainsi que l'aménagement de voies en site propre ou encore de parkings relais afin d'inciter nos concitoyens à limiter leur usage de la voiture.

la commission

d'alimentation en eau potable ou d'assainissement, afin de faire face à l'augmentation des coûts de l'énergie. L'article 14 de la loi de finances prévoit un dispositif de compensation

de réduire le trafic aérien pour favoriser, lorsque cela est possible, des modes de transport alternatifs. Les vols en jet privé, aux tarifs inabordables pour une grande majorité de la population et aux taux d'émanation de CO2 par personne

en projet de loi de finances rectificative pour 2022. Je propose d'aller au-delà en me référant strictement aux calculs du Gouvernement. Il s'agit d'une bonne occasion de conjuguer isolation acoustique et isolation thermique, qui ont un double impact environnemental,

Les travaux d'insonorisation des riverains des aéroports pâtissent de l'effondrement du rendement de la TNSA depuis le début de la crise sanitaire, ce qui n'est pas acceptable.

les incendies l'été dernier. Ces feux sont un drame pour les paysages, pour la biodiversité et, plus largement, pour l'environnement. Il nous faut repenser la reforestation afin de mieux prendre en compte le risque incendie, notamment en travaillant à une diversification des plantations. Notre amendement vise à dégager les moyens financiers d'un reboisement massif

comme cela a été rappelé par M. le rapporteur spécial, le Sénat a également voté lors des débats sur le projet de loi finances rectificative 100 millions d'euros supplémentaires, qui seront en partie consommés en 2023, au-delà de l'exercice 2022, avec 50 millions d'euros pour le réseau national non concédé et 50 millions d'euros qui transiteront par les collectivités locales. C'est un effort important,

par l'Ademe, à hauteur de 100 millions d'euros, afin de nous donner réellement les moyens d'atteindre nos objectifs de réduction et de recyclage des déchets. Il faut en effet rappeler que la loi Agec du 10 février 2020 fixe plusieurs objectifs, dont notamment celui de réduire de 15 % les déchets ménagers et de 5 % les déchets économiques ou encore de tendre vers 100 % de plastique recyclé en 2025. Si les moyens alloués au fonds économie circulaire sont en hausse de 46 millions d'euros dans le présent PLF, il faut néanmoins rappeler que cette augmentation était attendue, du fait de la quasi-extinction en 2023 des crédits accordés au titre du plan de relance. Le rapporteur pour avis à l'Assemblée nationale, Stéphane Delautrette, a ainsi estimé que ce budget restait trop limité pour espérer atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement en matière de réduction des déchets. le précise ainsi dans son rapport, l'Ademe indique que de nombreux projets identifiés ne pourront être pris en charge par le fonds. En conséquence, il paraît nécessaire d'abonder les crédits du fonds économie circulaire à hauteur de 100 millions d'euros. Quel est l'avis de

n° II-219 rectifié . Mme de Cidrac propose de garantir un montant minimum de 20 millions d'euros dédiés aux activités de réemploi au sein du budget pour 2023 du fonds économie circulaire piloté par l'Ademe. Cette enveloppe permettra de soutenir la création et le développement d'infrastructures dédiées (ESS) spécialistes du réemploi et de la réutilisation, ainsi que des réseaux qui animent et accompagnent ce développement, comme les recycleries, les ressourceries ou les cet amendement, il s'agit d'accorder des crédits supplémentaires à hauteur de 20 millions d'euros pour soutenir la filière, à savoir le développement et le fonctionnement des structures et des infrastructures dédiées au secteur économique et solidaire,

confié aux éco-organismes et aux producteurs en système individuel fonctionnent mal. En clair, les éco-organismes font preuve de mauvaise volonté. Dans ces conditions, les structures du réemploi solidaire ne peuvent compter sur ces fonds pour subvenir à leurs besoins de financement, d'où la proposition d'abonder le budget de l'Ademe dans ce sens de 20 millions d'euros.

Cet amendement vise à augmenter les moyens alloués à la prévention des risques technologiques et des pollutions, à hauteur de 62 millions d'euros, soit le doublement des moyens existants. Les accidents récents, que je ne citerai pas, montrent à l'évidence la nécessité de renforcer les moyens de surveillance des installations. Cet amendement a pour ambition de répondre aux questions formulées par la commission d'enquête du Sénat sur la préservation des sols de la pollution.

amendement vise à créer 100 ETP dédiés à l'inspection des sites classés, afin de tenir compte des conclusions de la commission d'enquête sénatoriale sur l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, Rouen, rendues le 2 juin 2020. Dans celui-ci, les deux rapporteures, Mmes Bonnefoy et Bonfanti-Dossat, ont déploré les manquements graves nuisant à l'efficacité des mécanismes de prévention des accidents industriels et ont formulé en conséquence un ensemble de recommandations pour une meilleure prise en compte des risques y afférents. Parmi leurs constats, il faut noter celui de l'inadéquation entre les moyens humains et les objectifs fixés pour une meilleure prévention des risques industriels. Cette réalité semble d'autant plus forte que, l'été dernier, un nouvel incendie s'est produit sur un site Seveso situé à Bergerac. En réponse, le Gouvernement avait annoncé la création de nombreux postes pour l'inspection des sites classés, afin d'atteindre un objectif d'augmentation de 50 % de leur nombre. Or le bilan semble aujourd'hui très en deçà des attentes et des besoins et seule une cinquantaine d'inspecteurs auraient été recrutés. Nous estimons qu'un effort important doit être consenti dès 2023, afin que certains drames ne se reproduisent pas. Nous proposons ainsi la création

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement porté par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable vise à sécuriser l'attribution de 15 millions d'euros au sujet de la prévention des inondations, dans le cadre du fonds vert, dont on ne connaît pas à ce jour la ventilation. Le risque inondation est le premier risque naturel auquel la France est exposée, compte tenu du nombre de communes concernées et des dommages qu'il peut provoquer. Depuis 1982, les deux tiers des indemnisations au titre des catastrophes naturelles ont été déclenchées à la suite d'inondations, pour un montant moyen d'environ 570 millions d'euros par an. Il est estimé qu'environ 17 millions d'habitants se situent en zone potentiellement inondable, ainsi que 40 % des emplois. Ces crédits ont vocation à constituer des crédits d'intervention et de transferts aux collectivités, pour un montant de 15 millions d'euros. gaz. Quel est l'avis de la commission ?

L'État n'ayant pas tenu cet engagement, le coût des investissements a été supporté par l'exploitant local, qui s'est trouvé contraint de le répercuter sur le prix du gaz, à hauteur de près de 4 euros par bouteille. C'est donc le consommateur martiniquais qui finance un investissement dont la responsabilité revenait au moins en partie à l'État. La consommation de gaz en bouteilles est largement répandue à la Martinique, en particulier dans les foyers les plus modestes. Les augmentations de prix ne sont plus soutenables pour un grand nombre de familles. Cet amendement vise donc à rétablir de l'équité au travers de la création d'un fonds qui permettra à l'État de prendre sa part dans les investissements, comme cela était prévu initialement, et de faire baisser d'autant le prix de la bouteille de gaz. Quel est l'avis de la commission ? La commission La commission n'a pas d'avis sur ce sujet extrêmement technique et précis, mais souhaite savoir si le Gouvernement a tenu ses engagements, tels qu'ils étaient prévus par la convention tripartite. Quel est

Malgré l'augmentation des crédits consacrés à l'entretien courant et préventif du réseau prévu par la loi de finances pour 2023, les montants prévus restent bien inférieurs aux besoins. Les documents budgétaires l'indiquent sans détour la dégradation de l'état des routes nationales se poursuit. La proportion des chaussées nécessitant un entretien de surface ou de structure devrait passer, monsieur le ministre, de 45,9 % en 2021 à 50 % en 2022. Alors que la loi 3DS prévoit la possibilité pour les départements, les métropoles et les régions intéressées de se voir transférer des portions de route du réseau national non concédé, il est crucial de s'assurer que l'État ne baisse pas la garde et investit suffisamment dans le réseau, à la veille de ces transferts. Sinon, cela provoquera bien sûr un mouvement de recul et une non-adhésion

il faut le reconnaître, les crédits que l'État consacre à l'entretien des routes nationales progressent, notamment grâce à l'augmentation des fonds de concours versés à l'Afit France. À la faveur de cette augmentation, ces crédits dépassent la trajectoire prévue par la LOM, qui était de 850 millions d'euros en 2022 et de 930 millions d'euros en 2023.

permettra de proposer une prime supplémentaire à l'achat ou au rétrofit de 1 000 camions électriques de plus de 5 tonnes. Il pourra ainsi inciter les transporteurs à s'équiper en camions électriques, dont le coût d'acquisition reste élevé. Quel se verra contrainte d'émettre un avis défavorable. En complément des dispositifs que j'ai cités tout à l'heure, qui visaient à la fois les camions et les bus, il existe un dispositif de suramortissement pour l'acquisition de véhicules lourds, lourds, prévu à l'article 39 A du code général des impôts, valable jusqu'en 2030. Dans le cadre de la première partie du PLF, nous avons déjà adopté plusieurs mesures en faveur des poids lourds, à savoir un prêt à taux zéro en faveur du verdissement des poids lourds, prévu à l'article 8 E, et une extension à la pratique du rétrofit du suramortissement que j'ai évoqué

15 millions d'euros supplémentaires à l'appel à projets « Écosystème des véhicules lourds électriques », ouvert en mars 2022 et doté de 65 millions d'euros.

tout ce qui a été évoqué au sujet de l'amendement précédent, à savoir le dispositif de suramortissement, le prêt à taux zéro du verdissement des poids lourds et une extension à la pratique du rétrofit du suramortissement.

à mettre en oeuvre les politiques de prévention des risques naturels majeurs, risques qui se multiplient et qui sont même appelés à devenir la norme dans les prochaines années, comme de nombreuses études scientifiques le démontrent. Le présent amendement prévoit donc d'établir à hauteur de 250 millions d'euros le montant des crédits alloués au fonds Barnier, soit une augmentation de 45 millions d'euros. Quel est l'avis de la commission

Dans ce contexte où le réchauffement climatique joue un rôle majeur, il est incompréhensible de réduire le budget de ce fonds, qui risque d'être sollicité davantage. Malheureusement, réponse a déjà été donnée

quand elles sont endommagées par une catastrophe naturelle- affaissement de terrain à la suite d'une inondation, rétractation de sol à la suite d'une sécheresse, apparition de cavités liée au réchauffement climatique, etc. Il est ainsi proposé de créer un nouveau programme « Fonds de réparation des infrastructures de transport non assurables », doté de 40 millions d'euros. Quel

fameuse raffinerie et des atteintes graves sur l'environnement et la santé publique qu'elle entraîne. Cet institut composé de citoyens, de volontaires, d'élus et de scientifiques a pour objet d'effectuer des relevés et des études de terrain publier ensuite ces données, d'organiser des débats et de sensibiliser tout un territoire sur des enjeux de santé environnementale. Cette démarche, fondée sur la démocratie participative, mais aussi l'expertise scientifique et une vigilance citoyenne, commence à faire des émules

fonds de 20 millions d'euros, qui viendra en appui des instituts écocitoyens dans un partenariat à définir. Quel est l'avis du Gouvernement ?

qu'il est souhaitable de détruire, notamment au travers d'une filière de recyclage. Cette ligne budgétaire offrira aux collectivités la possibilité de démanteler les navires hors d'usage dans la commune.

Denise Saint-Pé. Cet amendement vise à faciliter la recherche et le développement de la décarbonation des navires. L'Organisation maritime internationale a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre des navires d'au moins 50 % d'ici à 2050. Mis en place en 2022 et reconduit en 2023, le fonds d'intervention maritime (FIM) est notamment destiné à soutenir financièrement le développement d'activités maritimes durables, telles que le transport vert. Cet amendement s'inscrit dans cette logique, avec une dotation de 10 millions d'euros pour le FIM visant à développer la recherche sur la décarbonation des navires. La commission partage

Malgré leur situation insulaire, les territoires des Antilles, en particulier, sont confrontés à une importante crise du secteur de la pêche liée à plusieurs facteurs. Les comités sont, par ailleurs, amenés amenés à jouer un rôle d'accompagnement technique important dans le nécessaire renouvellement de la flotte, d'ailleurs soutenu par le Gouvernement, qui est l'un des éléments de réponse à la crise. Une aide exceptionnelle d'environ 200 000 euros par comité permettrait d'aider le secteur à se moderniser. C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à dégager une enveloppe globale de 1 million d'euros supplémentaires.

portant sur 50 % de l'encours du prêt, sous conditions de ressources, afin de soutenir les familles modestes souhaitant s'orienter vers des véhicules moins émetteurs, notamment hybrides rechargeables ou électriques. Quel

Si le fonds vert prend une teinte de bleu, je retire

Le plafond d'emplois de l'Ademe sera relevé de 90 équivalents temps plein en 2023. Le rehaussement de ce plafond d'emplois était nécessaire dans la mesure où, en 2022, l'agence a été contrainte de recruter des intérimaires pour faire face à l'élargissement de ses missions. Notre préoccupation est de renforcer l'offre d'ingénierie pour accompagner les collectivités dans la transition écologique. Il s'agit là d'un enjeu majeur auquel on ne pourra répondre sans moyens humains à la hauteur.

effectifs supplémentaires. Il importe de donner au Cerema des moyens humains et budgétaires à la hauteur des enjeux auxquels la population et les collectivités territoriales sont confrontées. L'amendement

du personnel au Cerema, qui est un partenaire des territoires en matière d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement et le changement climatique. Nous fonctionnons à moyens constants, c'est vrai.

Depuis 2013, il a perdu 734 ETP. C'est pourquoi cet amendement vise à augmenter ses effectifs, afin notamment de lui permettre d'assurer ses missions relatives à l'adaptation du territoire au changement climatique. À la suite d'un été particulièrement marqué par les feux de forêt et les vagues de chaleur successives, nous ne pouvons faire l'économie de crédits supplémentaires pour renforcer les moyens humains de cet opérateur.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

est vrai que cette enveloppe est gelée depuis des années, mais il s'agit d'une dotation d'investissement. Si vous abondez cette enveloppe, vous abondez

qui atteint désormais un niveau critique, mettant met en danger sa capacité à financer l'indemnisation de possibles contentieux qu'elle serait amenée à perdre. Il est donc indispensable, dans le contexte d'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire national de voyageurs,

sur le modèle de la brigade alpine, qui comprend 16 louvetiers, cet amendement vise à abonder de 2,5 millions d'euros le budget de l'Office français de la biodiversité, afin de permettre l'embauche d'une cinquantaine de louvetiers, à répartir dans les trois brigades supplémentaires qui

faire face au changement climatique et préserver la biodiversité. Or les dotations de fonctionnement représentent, en valeur cumulée, environ 1,3 million d'euros par an pour l'ensemble des conservatoires, soit 1 200 euros par ETP. Afin de maintenir les compétences indispensables des équipes et de faire face à l'évolution des charges en raison de l'inflation, le présent amendement vise à porter le budget du réseau à 3,5 millions d'euros en abondant l'action correspondante de 2,2 millions d'euros supplémentaires. L'amendement n° II-905 rectifié, qui

est à M. Hervé Gillé. Cet amendement vise à doter les conservatoires d'espaces naturels des moyens nécessaires à la bonne réalisation des missions qui leur sont confiées.

Aussi, cet amendement vise à abonder l'action n° 07 Gestion des milieux et biodiversité, du programme 113, « Paysage, eau et biodiversité », de 1,5 million d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

avec l'ambition affichée et les objectifs annoncés par le Gouvernement pour l'accompagnement de la stratégie nationale biodiversité 2030. Ce serait un signal politique fort à l'approche de la COP15 sur la biodiversité.

le rapporteur pour avis. Cet amendement de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable vise à augmenter de 270 000 euros les crédits de l'action n°

il est proposé de rehausser la trajectoire des emplois de l'ASN dès 2023, de façon relativement modeste- 270 000 euros pour trois postes -, y compris pour tenir compte du fait que les profils recherchés par l'Autorité constituent des métiers particulièrement en tension. l'avis de la commission ?

Cette ligne complémentaire doit permettre, d'une part, le déploiement des modalités de contrôle de la gestion de projets complexes comme les opérations de démantèlement ou la reprise et le conditionnement des déchets nucléaires ; d'autre part, le développement des expertises collectives menées par l'ASN en lien avec ses partenaires.

Je rappelle que le projet de loi de finances pour 2023 prévoit que les effectifs de l'ASN seront augmentés de 6 ETP, notamment pour renforcer le contrôle de la gestion des projets complexes et des expertises collectives. L'ASN fait par ailleurs appel aux expertises réalisées par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). La détermination par l'IRSN de la part de la subvention dévolue aux missions d'appui technique au profit de l'ASN fait l'objet d'une consultation préalable de cette dernière, sur le fondement de l'article L. 592-24 du code de l'environnement. De façon générale, le budget de l'ASN se trouve au sein d'un programme budgétaire beaucoup plus large, ce qui lui permet des redéploiements en cas de besoin. Il n'est donc pas nécessaire d'ouvrir des crédits complémentaires sur cette ligne.

Les crédits, on le sait, sont rattachés au programme 174, « Énergie, climat et après-mines ». Entre janvier et août 2022, 416 000 primes ont été attribuées. Si l'on ne tient compte c'est super ! Mais, dans les faits, le bilan est vraiment très faible en termes de gains d'efficacité énergétique. Un indicateur de performance a été rattaché au programme 362, « Écologie Écologie », de la mission « Plan de relance ». Il montre que, en 2021, sur un objectif de 80 000 logements, seuls 2 100 logements rénovés grâce à la prime de transition énergétique ont perdu le statut de passoire thermique, qui correspond aux étiquettes F ou G. Quel échec ! De manière un peu similaire, la Cour des comptes avait relevé dans un rapport de mars 2022 que seuls 2 500

monsieur le président

? Cet amendement est satisfait, puisque les agents et salariés qui occupent des logements de fonction peuvent bénéficier de MaPrimeRénov'sous conditions s'ils souhaitent réaliser des travaux de rénovation énergétique dans un autre logement qu'ils détiennent et qu'ils prévoient d'affecter à leur résidence principale à l'issue de leur activité. de leur activité. Les logements éligibles incluent ceux qui sont occupés à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires de droits réels immobiliers dans un délai maximum d'un an suivant la demande du solde de la prime.

Il est nécessaire de créer les conditions d'application d'une véritable contribution écologique du transport routier de marchandises, selon le principe « pollueur : payeur ». Cela favorisera la transition énergétique et le report modal. Depuis plusieurs années, nous ne cessons de proposer que les entreprises qui décident du transport, les donneurs d'ordres, soient redevables d'une écocontribution visant à la réalisation des objectifs inscrits dans la loi d'orientation des mobilités. Cette écocontribution serait pédagogique pour les donneurs d'ordres, pérenne pour le financement, l'entretien et la rénovation des infrastructures, et permettrait de toucher le trafic européen qui a pour origine ou destination la France. Sa mise en place utiliserait un dispositif existant depuis le Grenelle de l'environnement, qu'il suffit d'appliquer, donnant un coût à la tonne de CO2 déclarée aux donneurs d'ordres par les transporteurs.

qui pourraient être collectés pour financer la transition des routes, des flottes et du report modal. Nous souhaitons qu'une partie de ce rapport soit consacrée au dispositif de taxe de valorisation environnementale (TVE), développé depuis plusieurs années par Philippe Mangeart, et qu'il semblerait pertinent d'expérimenter. se basant sur la volumétrie carbone que les transporteurs communiquent à leurs clients pour chaque opération, il serait simple de calculer la contribution de ces derniers à l'utilisation des infrastructures. Pour cela, ce rapport serait particulièrement utile.

à coût constant, selon les déclarations du Gouvernement, le dispositif d'amortisseur ; et d'anticiper les versements de compensations dus aux fournisseurs d'électricité au titre des dispositifs de bouclier et d'amortisseur. Madame la ministre, nous avons de très nombreuses questions, qui restent en suspens malgré les éléments que vous nous avez communiqués hier et ce matin. Ces questions portent aussi bien sur le bouclier que sur l'amortisseur, puisqu'un certain nombre de dispositions ont été annoncées par voie de presse, voire sur d'autres supports de communication, mais que le dispositif législatif

paraissent fondamentaux. Nous aimerions, madame la ministre, que vous indiquiez au Parlement le nombre d'éligibles pour le bouclier sur le gaz et l'électricité, par catégorie d'entités, notamment s'agissant des collectivités territoriales et des petites entreprises, ainsi que le volume de consommation d'électricité ouvert.

les caractéristiques du dispositif en faveur du chauffage collectif électrique que le Gouvernement a annoncé vouloir mettre en oeuvre par décret ? Sera-t-il aussi protecteur que le bouclier ?

que vous nous confirmiez formellement, ici, devant le Parlement, la liste de toutes les entités qui seront éligibles au mécanisme. L'ensemble des paramètres structurants du dispositif sont également renvoyés à un décret. Des annonces ont été faites le 29 novembre dernier, mais, là aussi, nous demandons que Mme la ministre prenne des engagements formels sur la définition de ces paramètres. En effet, dans le PLF

que tous les consommateurs seront soumis au même dispositif d'amortisseur ? L'article prévoit aussi que le dispositif d'amortisseur soit suspendu en cas de délestage.

Mme la ministre.

au champ des ETI et des grandes entreprises pour faciliter le travail des fournisseurs d'électricité. Aujourd'hui, les grands fournisseurs nous annoncent pouvoir appliquer ce dispositif sur la facture dès la fin du mois de janvier.

à la marge les dispositions présentées à l'Assemblée nationale. Il prévoit tout d'abord une simplification du dispositif « amortisseur électricité » afin que la réduction de prix dont bénéficie chaque client soit calculée sur la base du prix de l'électricité figurant dans son

de limiter considérablement notre consommation, de même que les baisses de tension ou les contrats d'effacement et d'interruptibilité qui ont été négociés. Toutes ces mesures seront activées avant de passer à la mesure de protection ultime pour éviter le black-out. Dans une